J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires est parvenue à l'adoption d'un texte commun.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la crise sanitaire a montré, s'il en était encore besoin, que les États, loin d'être obsolètes, pouvaient beaucoup. En outre, elle a montré la nécessité et l'efficacité de la politique budgétaire, quand cette dernière n'est pas paralysée par des contraintes arbitraires. En France, comme dans la plupart des pays avancés, les finances publiques ont pris en charge une grande partie des dépenses à la suite de la chute du PIB. L'explosion du chômage ou les faillites en chaîne ont ainsi été évitées. Les taux d'intérêt sont restés négatifs pour les échéances inférieures à dix ans et faibles pour les échéances à long terme. À l'avenir, les nécessités de la transition écologique imposeront une forte hausse des investissements publics. Depuis des années, la social-démocratie n'a de cesse de prôner un rationnement de la puissance publique au service

Malgré tout, en France, d'aucuns s'interrogent : la gauche réformiste a-t-elle encore un avenir ? Comme Mark Twain lisant le faire-part de son décès dans un journal, elle répondra : « L'annonce de ma mort est très exagérée. » Il est vrai qu'elle en a vu d'autres depuis le congrès de Tours, il y a un siècle ! y a un siècle ! Ce Lazare social-démocrate est toujours ressuscité pour continuer son oeuvre de réforme. Ceux qui doutent de cette résilience liront l'essai précis et alerte d'Henri Weber, qui a siégé sur ces travées - je souhaite rendre hommage à ce grand acteur et analyste de la social-démocratie française. Conciliant avec obstination socialisme et liberté, sûre que le libéralisme produit avant tout de l'injustice tandis que le communisme conduit à la tyrannie d'une minorité, l'inénarrable social-démocratie a connu trois époques depuis la guerre. D'abord celle de la conquête. Pendant la période de croissance rapide appelée les Trente Glorieuses, elle a mis en oeuvre l'essentiel des réformes qui constituaient la trame des revendications ouvrières Je pense notamment à la protection générale contre les aléas de la vie, à la régulation du marché du travail, à l'extension des congés payés, au droit syndical, au pilotage keynésien de l'économie, toutes ces réformes transformant radicalement la condition salariale dans les pays développés. social-démocratie se tourna vers des compromis défensifs, destinés autant à maintenir les acquis de la période précédente qu'à contenir les effets délétères de la faible croissance et du chômage de masse. masse. Pour aborder la faculté de la social-démocratie à faire évoluer notre pays, nul besoin d'aller chercher dans l'Histoire des dates trop lointaines. Il y a plus de sept ans, nous engagions des réformes sociales sans plomber les comptes publics. D'ailleurs, si l'on compare la situation d'aujourd'hui à celle qu'a laissée Nicolas Sarkozy

François Hollande a été celui qui aura fait sortir la France de la procédure disciplinaire pour dérapage budgétaire lancée par Bruxelles en 2009. Néanmoins, cela n'a pas empêché des idées radicales d'occuper le débat public. Pour certains, il suffit d'interdire les déficits, par la loi ou, mieux encore, par la Constitution ! De prime abord, nous pourrions penser qu'une telle décision aurait pour vertu de convaincre les investisseurs et les marchés financiers de l'irréversibilité de la conversion des États européens à la discipline budgétaire, et, ce faisant, de restaurer leur confiance. Le problème, c'est que ce raisonnement ne résiste guère à l'expérience. Tout d'abord, il ne suffit pas de promulguer des textes de loi pour transformer la réalité. De nombreuses règles contraignantes en matière budgétaire en Europe existent déjà, sans que cela ait nullement empêché les États de creuser leurs déficits et d'augmenter leur dette. Prôner la règle d'or selon laquelle l'évolution des dépenses publiques doit être inférieure à celle des recettes, tout en écartant des modifications du taux des prélèvements obligatoires, comme l'a proposé la commission Arthuis, est encore pire cela revient à empêcher toute politique budgétaire de soutien à l'économie. À l'avenir, la dépense publique doit aussi être mobilisée à plus long terme, puisque la France doit réaliser la transition écologique et favoriser le redéploiement des services publics

Le problème vient de la dégradation, faute de moyens, de ces derniers, qui est source d'inégalités sociales et territoriales importantes. C'est là toute la différence entre les sociaux-démocrates et les sociaux-libéraux. Mais l'heure n'est plus aux sociaux-démocrates dans ce pays. Le parfum ambiant respire le libéralisme décomplexé, et les choix budgétaires de ces dernières années

pour être à l'équilibre ne me semble pas être une politique budgétaire dessinant un cap digne de ce nom. La gestion comptable et austéritaire des comptes publics ne peut constituer à elle seule l'horizon indépassable des réformes.

au milieu du XIX siècle, le député Frédéric Bastiat affirmait qu'il n'y a rien de plus facile que de voter une dépense, et rien de plus difficile que de voter une recette. De prime abord, le bilan de l'examen du projet de loi de finances pour 2022 au Sénat semble lui donner tort, puisque la Haute Assemblée a voté toutes les recettes du budget, ... et aucune dépense. Mais je crois que nous avons, en fait, confirmé la maxime de Bastiat.

de cibler les dépenses à couper pour réduire effectivement le déficit public. Il a préféré rejeter en bloc le budget pour 2022. Tel est donc l'exercice auquel nous sommes invités aujourd'hui : critiquer en bloc, pour ne pas discuter dans les détails. Je doute que le fait de verser dans des considérations générales et abstraites, plutôt que de procéder à l'examen des différentes missions, serve notre institution. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire la semaine dernière, notre groupe regrette profondément cette décision. Nous aurions préféré mener les discussions budgétaires jusqu'à leur terme. La critique est aisée, l'art est difficile. Ce sont vos mots, monsieur le rapporteur général. Quelle crédibilité avons-nous encore sur l'impératif de réduction des dépenses publiques, alors que nous avons renoncé à notre pouvoir, voire à notre devoir, de voter les dépenses ? Néanmoins, le sujet est trop grave pour que nous nous refusions à confronter nos points de vue. Je vais donc tâcher de dresser un bref diagnostic et d'esquisser quelques pistes de solutions. Jamais, en temps de paix, notre pays n'a été aussi endetté.

le ratio d'endettement était le même en France et en Allemagne, autour de 65 % du PIB. Aujourd'hui, le ratio français a augmenté de 50 points et s'élève à 115 %, quand celui de nos voisins allemands est Cette situation est très préoccupante. Bien sûr, les crises sanitaire et financière expliquent pour une large part l'explosion de notre dette, mais l'Allemagne, qui a connu les mêmes crises, s'en sort beaucoup mieux. Il y a donc un mal français qui nous empêche de réduire notre dette, qui fragilise la situation de nos comptes publics et qui menace notre souveraineté nationale : ce mal français, c'est notre immense difficulté à réduire la dépense publique et à réformer l'État. Certains, ici, pensent que le Gouvernement actuel en porte toute la responsabilité. Certes, les dépenses publiques n'ont cessé de croître au cours du quinquennat, mais il est également vrai que ce gouvernement est le seul à être parvenu, au cours des quinze dernières années, à stabiliser la dette publique. Avant la crise sanitaire, le déficit était maîtrisé et le taux d'endettement avait même commencé de baisser. Ainsi, en l'occurrence, il est trop facile de critiquer le Gouvernement sur son impuissance à faire baisser la dépense publique, sans jamais indiquer quelles dépenses il aurait fallu réduire. Voilà, à mes yeux, la cause profonde de ce mal français, qui nous empêche de réduire notre dette publique. J'ai cru utile de remettre ainsi les pendules à l'heure, car nous devons, sur ce sujet, tenir un discours de vérité. Il est trop facile de prêcher sans cesse la réduction des dépenses publiques sans jamais se risquer à préciser le propos. au cours de la crise sanitaire, le Sénat a voté tous les projets de loi de finances rectificative, exception faite du tout dernier. Il est donc aisé de dénoncer aujourd'hui la hausse des dépenses publiques, alors que nous avons soutenu, je vous le rappelle, mes chers collègues, le « quoi qu'il en coûte C'est d'autant plus grave que, pour relever les défis auxquels notre pays fait face, au premier rang desquels se trouvent la transition écologique et la révolution numérique, la puissance publique devra jouer un rôle majeur de soutien à l'innovation. Ainsi, le plan France 2030, présenté par le Président de la République, a fixé des objectifs ambitieux d'investissement public dans des verticales clefs de rupture technologique. Ces injonctions sont apparemment contradictoires : d'une part, nous devons nécessairement réduire les dépenses publiques, pour abaisser notre endettement ; d'autre part, nous devons poursuivre l'investissement public, afin de ne pas décrocher, dans tous les domaines stratégiques, notre souveraineté nationale et notre capacité à créer de la valeur. Je suis convaincue, mes chers collègues, que nous avons tous à coeur de relever cet immense défi. Bien sûr, nos sensibilités politiques et nos différences d'approche nous opposeront sur les chemins à emprunter pour y parvenir, mais il nous faudra bien accepter, le moment venu, de remettre sur le métier

le budget pour 2022, que nous venons de rejeter, ne fait qu'accentuer les risques pesant sur la soutenabilité de nos finances publiques pour l'avenir. Depuis 2017 et jusqu'au début de la crise sanitaire, le Sénat a rappelé régulièrement au Gouvernement la nécessité d'assainir les comptes publics tant que la croissance économique le permettait, compte tenu du niveau de déficit et d'endettement de nos administrations publiques,

une phrase de John Fitzgerald Kennedy : « Le meilleur temps pour réparer sa toiture, c'est lorsque le soleil brille. » Malheureusement, comme souvent, le Sénat n'a pas été entendu et, lorsque la tempête s'est abattue sur l'économie mondiale

%. Certes- il faut s'en réjouir -, l'embellie économique a été particulièrement marquée en France au cours des derniers mois, entraînant un

alors que les nouvelles émissions de dette vont encore représenter 260 milliards d'euros dans le budget de l'État ... Au contraire, les recettes tirées de ce regain inattendu de croissance auraient pu et auraient dû être employées à réduire

de voir ce qu'il est advenu des travaux d'Action publique 2022 ou de considérer l'absence totale de réflexion sur la relance de la décentralisation, alors que les Français plébiscitent les actions de proximité menées par les collectivités locales durant la crise, notamment par les communes. qu'en est-il pour l'avenir ? Il ne suffit pas de marteler, comme le fait Bruno Le Maire dans les médias, que « tout va bien », que l'économie repart et que l'on est parfaitement rassuré sur l'état de nos finances publiques !

le secrétaire d'État, quel est votre plan ? Quelle est la stratégie du Gouvernement ? Quelles sont les réformes qui pourraient vous permettre de tenir, cette fois-ci, votre objectif

avec des versements d'argent public, sans contrôle et sans capacité d'action réelle. Il faut réhabiliter la dépense publique, mais non pas cette dépense-ci, qui est injuste.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je vais vous parler de la réforme de l'État, même si cela n'a pas l'air de passionner grand monde ce soir ... Les débats relatifs à la réforme de l'État ont pour seule et unique finalité l'assainissement des comptes publics- c'est toujours vrai aujourd'hui -, comme si une réforme étatique ne pouvait être autre chose qu'une optimisation des coûts. Jean Rostand écrivait d'ailleurs : « Les mauvais effets d'une juste réforme ne condamnent point cette réforme, mais la société. Certes, il faut équilibrer les comptes de l'État, mais nous restons persuadés que cet unique objectif dévitalise la société dans ses rapports avec l'administration. Nous sommes las de ce discours réformateur, politiquement mobilisateur et électoralement rentable.

Les fonctionnaires y ont vu, très majoritairement, un affaiblissement de l'État au bénéfice du secteur privé et une atteinte aux valeurs du service public ; en outre, les méthodes appliquées ont semblé arbitraires ou simplistes.

s'engager dans la modernisation, tendre vers la simplification et, pour finir, concrétiser la proximité. Emmanuel Macron, chef de projet, affirmait : « La mise en oeuvre des réformes que nous préconisons permettra d'améliorer les comptes publics d'une trentaine de milliards d'euros à l'horizon 2022. Ces réformes auraient été justifiées par la demande des Français : amélioration de l'information et de l'accueil des usagers, simplification des procédures, développement des échanges électroniques- je pense que M. le secrétaire d'État en parlera -, mais comment répondre à ces aspirations si ce n'est avec un État moins centralisé, la prise d'initiative et de responsabilité serait davantage valorisée et l'agent aurait des droits nouveaux d'intervention ? Les fonctionnaires seraient « trop nombreux ». Tous les libéraux font campagne sur la réduction

« nouveau monde » avec, une fois n'est pas coutume, de l'« ancien », avec l'annonce de la suppression de 120 000 emplois publics, dont 50 000 dans la fonction publique d'État, et on nous ressort les recettes de la RGPP avec la réforme de la rémunération des agents publics. Pour ce gouvernement, la modernisation et la simplification de la relation entre État et usagers sont d'ailleurs associées au tout-numérique. Cette perspective constitue un basculement

L'objectif est clair : inventer des « services publics sans administration, auto-organisés par des communautés de citoyens prenant leur part de leur opération par leurs contributions et leurs interactions » écrivait Henri Verdier, directeur interministériel du numérique et du système d'information et de communication de l'État. Le Conseil d'État a quant à lui évoqué « les conséquences disruptives pour le service public de l'émergence des plateformes numériques qui le concurrencent directement ». Mes chers collègues, la réforme de l'État doit-elle forcément s'inspirer des méthodes du privé ? Le président veut « plateformiser » l'État, ce qui n'est pas étonnant : cela permet de minimiser les responsabilités d'un donneur d'ordre, de transférer les risques aux travailleurs et une partie des prérogatives des employeurs aux usagers. un coup triple pour le libéralisme, qui veut réduire les coûts, s'affranchir de ses responsabilités et achever de transformer le citoyen en client. Une telle idée de la réforme contribue à saper l'État et le travail des fonctionnaires, qui sont confrontés à une perte de sens et d'expertise, le tout sans bénéfices pour les comptes publics.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je vous dis clairement, le groupe Union Centriste aurait bien entendu préféré que l'on puisse examiner

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la crise structurelle que connaît notre système de santé depuis plusieurs années a été aggravée par la crise conjoncturelle de la covid-19. de la covid-19. Elle a mis en lumière ce que soignants et élus dénonçaient depuis déjà trop longtemps : malgré les réformes successives engagées, nous faisons face à la nécessité d'une transformation en profondeur de notre système de soins. sociale) pour 2022 a été l'occasion de constater, pour la deuxième année consécutive, une aggravation sans précédent des comptes de la sécurité sociale. Celle-ci a enregistré en 2020 le plus lourd- et de loin -déficit de son histoire : il atteint près de 40 milliards d'euros sur l'ensemble des régimes obligatoires de base. C'est 10 milliards d'euros de plus que le précédent record, qui datait de 2010, au plus fort de la crise financière qui avait débuté en 2008. Et pour cause ! La crise de la covid a engendré une perte colossale des recettes, accompagnée d'une augmentation tout aussi colossale des dépenses de santé. Le déficit sera encore de 35 milliards d'euros cette année, et devrait malheureusement se pérenniser à un niveau très élevé. L'État a joué son rôle d'amortisseur et de protecteur durant la crise. Il était impensable de ne pas agir en conséquence, même si cela signifiait que le retour à l'équilibre des comptes sociaux s'éloignait durablement. Le « quoi qu'il en coûte » a été salutaire, et il n'est pas question ici de le remettre en cause. Néanmoins, notre rôle de législateur, mais aussi d'élus locaux et, pour ma part, de médecin nous engage à voir plus loin : il faut reconstruire dès aujourd'hui une trajectoire de retour à l'équilibre des comptes sociaux. Pour ce faire, la mesure de l'ampleur des déséquilibres actuels. Les dépenses de l'assurance maladie ne sont pas, comme dans le budget général de l'État, des dépenses d'investissement : il s'agit de dépenses de répartition, qui doivent donc être équilibrées. C'est pourquoi la Cades, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, financée par un impôt spécifique, a été créée pour rembourser la dette de la sécurité sociale. Or, en 2021, pour 1 000 euros dépensés dans la branche maladie, 130 euros sont financés par de nouvelles dettes à la charge des générations futures. Nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une telle situation,

Bien qu'indispensables et urgentes, elles représentent près de 40 % des dépenses supplémentaires en 2022. Enfin, les nouveaux traitements, plus ciblés et plus innovants, coûtent naturellement beaucoup plus cher. Sur ces sujets, il est impensable de revenir en arrière la France doit permettre à tous les patients d'accéder au meilleur traitement et aux soignants de travailler dans les meilleures conditions. Il faudra donc faire des économies, mais pas en matière de qualité des soins et pas n'importe comment. Dans un premier temps, il nous faut mieux évaluer nos politiques de santé. Cela passe par un PLFSS réformé, comme nous l'avons voté il y a quelques semaines. Cela passe aussi, de l'avis général du Sénat, par un recentrage de la sécurité sociale sur ses missions premières. Ainsi, le transfert, en 2020, de Santé publique France à l'assurance maladie a a considérablement plombé les comptes de la sécurité sociale. Il n'est pas normal que l'État ne compense pas ce transfert à son coût réel, mettant encore plus en difficulté les comptes sociaux. Dans un second temps, il faut sans doute lutter davantage contre la fraude, car il n'y a pas de petites économies. La gestion des dépenses doit aussi passer par un effort sur la réduction des soins redondants, des soins, leur gradation en fonction des besoins individuels, la généralisation du dossier médical partagé et la facilitation du maintien à domicile. Enfin, les recettes de la sécurité sociale ne peuvent plus reposer exclusivement sur le travail. Il nous faudra inventer d'autres sources de financement, sans quoi chaque nouvelle crise fera de nouveau plonger durablement nos comptes sociaux dans le rouge. Nous avons besoin d'un financement pérenne pour que cette instabilité cesse de peser comme une menace sur notre système de soins, et pour ne pas transmettre cette charge aux futures générations. Nous avons beaucoup entendu parler du projet de « grande sécu », notamment par la voix du ministre de la santé, qui teste sans doute ce sujet en vue de la campagne L'idée est lancée, le débat est ouvert. Il s'agit d'une prise en charge intégrale par l'assurance maladie obligatoire d'un panier de soins aux prix encadrés. Les complémentaires seraient cantonnées à rembourser les actes médicaux aux tarifs libres ou, par exemple, les frais de chambre individuelle.

Je n'ai pas de solution toute trouvée, mais j'ai la conviction qu'un tel débat est indispensable. À l'aube de l'élection présidentielle, une refonte plus structurelle et plus durable est à construire.

budgétaires, à la différence des époques antérieures, où la réduction du nombre des fonctionnaires se fondait sur une vision selon laquelle l'État n'avait pas à intervenir dans l'éducation, le social ou l'économie. Ainsi, la stratégie de réduction ne s'accompagne plus d'une volonté de repenser l'action de l'État.

Conseil d'État : « Il nous faut ainsi revenir aux sources de l'intérêt général, qui n'est pas un mot creux, mais le ciment de notre société. Les hauts fonctionnaires doivent contribuer à le promouvoir, mais aussi à l'actualiser et à hiérarchiser les actions qui s'y rattachent. C'est un devoir qui s'impose à eux, même si le dernier mot ne saurait leur appartenir. » Il poursuit : « Il nous faut mieux conjuguer le court et le long terme et constamment relier l'action immédiate à une vision prospective et stratégique des politiques à conduire. Les exigences de l'action ne sauraient conduire à négliger les enjeux de moyen et long terme. Si les hauts fonctionnaires l'oublient, qui s'en chargera ? » Je me limiterai à la citation de ces mots puissants pour évoquer la réforme de la haute fonction publique, sur laquelle le Sénat a déjà largement exprimé son mécontentement, tant sur la forme que sur le fond. Réformer la haute fonction publique sans s'attaquer aux 483 taxes, impôts et cotisations, aux 3 500 pages du code du travail et aux 400 000 normes revient à donner un coup d'épée dans l'eau.

dressait le constat fort juste que « le numérique [ ...] permet de remplir conjointement [les] deux objectifs [d'un meilleur service public et d'une diminution des dépenses de fonctionnement] et c'est ce qui change [ ...] par rapport aux exercices précédents de réforme de l'action publique

sauf exception, l'occasion qui était offerte de repenser la politique publique ou la manière dont elle est administrée n'a pas été saisie. Un seul exemple : essayez de faire une demande de carte grise en France et faites de même en Finlande ... Vous constaterez par vous-même ! La simplification et la lisibilité ne sont pas les maîtres mots de la gouvernance de la politique du numérique.

Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, service numérique de la direction générale des entreprises, ambassadeur pour le numérique. Il me semble donc qu'il est possible, dans ce secteur, de gagner en efficacité et en efficience. Trois grands chantiers restent ouverts. L'inclusion numérique, tout d'abord, est largement perfectible. En la matière, la France a même rétrogradé,

souverain. Le 18 octobre dernier, plusieurs start-up françaises ont décidé de lancer leur propre initiative, contredisant le Président de la République qui, lors de la présentation du plan France 2030, estimait impossible pour la France de se doter d'un totalement souverain d'ici cinq ans.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, « figer l'État, c'est supprimer l'espérance, c'est supprimer l'action. [ ...] Si l'on se risquait à caractériser l'État d'aujourd'hui, on ne le pourrait qu'en introduisant [ ...] l'idée de mouvement

De surcroît, comme le souligne justement Jaurès, réformer est un mouvement permanent ; cela prend du temps. Nous constatons actuellement les conséquences néfastes de réformes brutales conduites dans le seul but de réduire la dépense publique.

Cette réforme, qui a opéré des réductions massives d'emplois publics à force de réorganisations de différents services, n'a pas pour autant redéfini les missions de l'État ni empêché la dépense publique de continuer d'augmenter. Est-ce à dire qu'il ne faut pas réformer l'État ? Absolument pas ! Les services publics doivent nécessairement s'adapter pour répondre aux besoins de la population. Ces dernières années, en effet, tout a changé. Grâce à l'informatique, de nouveaux services de démarches en ligne simplifient les demandes administratives des usagers. Il en est ainsi de la dématérialisation des titres sous l'égide de l'Agence nationale des titres sécurisés. Cette évolution, quoique souhaitable, doit néanmoins s'assortir de moyens humains. Les systèmes d'information et les logiciels nous permettent de gagner un temps précieux dans nos démarches. Cependant, nous devons faire en sorte qu'ils restent des outils au service des citoyens et des agents du service public, afin d'éviter que bon nombre

pour pallier la fermeture de nombreux services publics, les trésoreries notamment, peine encore à répondre aux besoins des élus et des populations. Si ces structures permettent d'accéder à certaines démarches administratives, l'accompagnement humain n'est pas à la hauteur des enjeux. Les écrans et les systèmes d'information, censés faciliter les démarches des citoyens, s'apparentent parfois à des barrières numériques. Garantir l'accès aux services publics de proximité, c'est lutter contre la fracture numérique, c'est renforcer le maillage territorial, c'est préserver la présence d'agents sur le terrain. Et c'est surtout s'en donner les moyens ! Réformer pour réformer, sans définir clairement les enjeux,

je vous remercie de vos interventions sur un sujet qui est évidemment au coeur des préoccupations des Français. Je tiens à excuser l'absence du ministre Olivier Dussopt, qui est en déplacement à l'étranger.

Cette gestion sérieuse nous a permis de faire baisser les impôts des Français et des entreprises : nous avons ramené le taux de prélèvements obligatoires à un niveau que nous n'avions pas connu depuis plus de vingt ans. Grâce à ces bons résultats, nous avons réussi à soutenir massivement notre économie, notamment pendant la crise.

Le scénario macroéconomique modifié sur cette base, les recettes de l'État s'en trouveront mécaniquement accrues, pour l'exercice 2021 comme pour l'exercice 2022. Il y a là autant d'indices qui viennent confirmer l'efficacité de la politique de soutien et de relance du Gouvernement et notre capacité à rétablir l'équilibre de nos comptes publics.

De même, nous estimions, au printemps dernier, que notre dette atteindrait 117,8 % du PIB en 2021 et 116,3 % en 2022 elle sera plutôt, en définitive, de 115,3 % du PIB en 2021 et de 113,5 % en 2022. Ces chiffres confirment ce que nous avons toujours dit depuis le début de la crise : c'est avant tout par la croissance que nous parviendrons à maîtriser nos comptes publics. ! Outre ces réussites en matière de conjoncture économique, l'année 2021 est aussi celle de la maîtrise et de la normalisation budgétaires. Nous avons en premier lieu annulé, pour 2021, les excédents de crédits mobilisés pour financer des besoins apparus au cours de l'année, notamment du fait de l'utilisation de la réserve de précaution. finances rectificative, plus de 2 milliards d'euros de crédits de la mission « Plan d'urgence face à la crise sanitaire », conformément à notre calendrier de sortie progressive des aides d'urgence. C'est une bonne nouvelle, qui laisse présager que bientôt nous laisserons la crise loin derrière nous et que 2021 sonne la fin du « quoi qu'il en coûte Deuxièmement, l'exécution des dépenses sur les budgets ordinaires des ministères en 2021 sera conforme au niveau prévu en loi de finances initiale, à l'exception de quelques compensations de pertes de recettes liées à la crise sanitaire et de la mise en oeuvre de l'indemnité inflation. Le

La maîtrise de nos comptes publics passe aussi par des outils renouvelés. J'aimerais à cet égard revenir sur la proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, que vous avez récemment adoptée. Vous vous êtes en effet entendus avec les députés sur ce texte proposé par Laurent Saint-Martin et Éric Woerth instituant un encadrement pluriannuel de la dépense publique. contient me semblent aller tout à fait dans le sens d'une meilleure maîtrise des dépenses publiques, dont la visibilité de long terme est une des composantes. Je souhaite par ailleurs revenir sur la réforme de l'État

Cette transformation s'inscrit dans une perspective claire : construire l'État de demain, celui d'une action publique plus proche, plus simple et plus efficace. Réformer l'État, tout d'abord, c'est répondre sans ambiguïté à la question de son utilité et de son impact. L'État n'est pas une machine bureaucratique tournée sur elle-même, sur ses fonctionnaires et sur les normes qu'ils édictent. L'action publique a pour moteur les conséquences concrètes qu'elle a sur la vie des Français. Au-delà de l'indispensable transparence, que nous avons renforcée le baromètre des résultats de l'action publique en ligne sur le site du Gouvernement,

d'une transformation plus profonde qu'une simple réforme organisationnelle de l'État ou qu'un exercice de révision générale des politiques publiques, comptables et budgétaires. Cette transformation, ensuite, c'est la réforme de l'État territorial, qui rapproche l'État des citoyens et renforce les moyens des territoires pour des réponses adaptées aux besoins de chacun. Dans cette transformation, le préfet occupe bien sûr- vous le savez mieux que quiconque -une place centrale : il est celui qui pilote une action interministérielle unifiée et cohérente et une vision stratégique du territoire appuyée et renforcée par l'expertise nationale. Nous avons pour la première fois instauré une feuille de route interministérielle pour chaque préfet de département et chaque préfet de région, signée par le Premier ministre, coconstruite avec chaque préfet et avec l'ensemble des services de l'État. C'est là une réelle responsabilisation des services déconcentrés. En contrepartie de cette responsabilisation, nous avons engagé un réarmement de l'État territorial en lui offrant davantage de compétences, d'expertise et d'ingénierie, ainsi que des marges de manoeuvre en matière budgétaire et de ressources humaines. Ce gouvernement met par ailleurs fin- enfin ! -à douze années d'appauvrissement de nos services déconcentrés au profit de nos administrations centrales. Nous faisons basculer le pouvoir de décision et les ressources au plus près du terrain, jusqu'à l'application de la norme. C'est à cette fin que nous avons autorisé les préfets à déroger à une norme nationale pour exercer leurs compétences au niveau local. a là, au sens propre, une révolution de l'action publique, qui sera désormais moins tournée vers la norme et davantage vers le résultat. Moins centralisée et plus proche du terrain, elle devient plus ouverte sur la société, plus bienveillante, accessible.

Quant à la réforme de la haute fonction publique portée par Amélie de Montchalin, elle contribue profondément à rebattre les cartes. Cette réforme doit refonder la formation, la carrière, le métier des hauts fonctionnaires ; on partira désormais d'une expérience opérationnelle et territoriale avant de construire des normes et des orientations nationales depuis d'une culture commune entre administrateurs, forces de sécurité, militaires, magistrats, hospitaliers. Bref, il s'agit d'une réforme ambitieuse qui participe pleinement de la transformation de l'action publique au bénéfice de l'ensemble de nos concitoyens. Nous allons

Monsieur le secrétaire d'État, si la présence de l'État en zone rurale est essentielle pour garantir à nos concitoyens l'accès aux services publics, la mise en oeuvre de cette présence au travers de l'organisation territoriale de l'État n'en pose pas moins question. La création des maisons labellisées France Services permet de conserver un accès aux services publics. Il faut cependant rappeler que ces structures sont essentiellement portées, aux deux tiers, par les collectivités territoriales et par d'autres acteurs tels que La Poste.

Pourtant, l'ambition initiale du Gouvernement était de couvrir tous les cantons à l'horizon de 2022. Force est de constater que pour le moment le compte n'y est pas, en ce qui concerne notamment la transformation prévue d'une centaine de sous-préfectures en maisons France Services. actuelle, seules 21 sous-préfectures sont labellisées et 13 en cours de labellisation. J'ajoute qu'était prévu également le financement de deux emplois permanents par maison. Là encore, l'État n'y met pas les moyens nécessaires : avec la dotation annuelle de 30 000 euros allouée au fonctionnement de chaque maison France Services, on est loin du compte. La crise sanitaire a mis en lumière, si besoin en était, la nécessité de réaffirmer la présence forte de l'État aux côtés des collectivités territoriales. Au-delà des engagements pris en la matière, l'État compte-t-il se donner les moyens de répondre aux besoins et aux enjeux de présence des services publics dans les territoires ruraux ?

pour la réplique. J'entends bien, monsieur le secrétaire d'État. Néanmoins, sur cet aspect des choses, l'État avait pris des engagements, notamment sur les sous-préfectures et sur l'accompagnement financier.

chacun comprend bien que, le jour où il y a un problème, il est beaucoup plus simple d'aller discuter avec une banque ou un groupe d'assurances français qu'avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde ! Monsieur le secrétaire d'État, le Gouvernement a-t-il une stratégie en la matière ?

nous. Demain, nous nous ferons dicter la loi. C'est déjà le cas d'ailleurs : quand nous avons négocié la dette européenne, l'Allemagne a commencé à nous dire qu'il fallait réformer nos retraites

et s'intensifie, le foisonnement des dispositifs à destination de nos entreprises nuit gravement à la lisibilité de l'action des pouvoirs publics. Or, résorber une partie du déficit, c'est aussi, nous semble-t-il, faire un exercice de transparence et de rationalisation du maquis fiscal des aides attribuées à nos entreprises, qui a considérablement gonflé, et sans contreparties, dans le contexte de la crise de

Avez-vous également prévu une réforme des aides versées aux entreprises pour mettre fin à ce véritable maquis fiscal ? Le « quoi qu'il en coûte » sera-t-il, à terme, uniquement payé par les salariés et les catégories les plus modestes ? À défaut, la moindre des choses serait de faire régner la transparence sur l'identité des entreprises bénéficiaires et les montants de crédits publics qui leur sont accordés.

qu'après cinq ans de macronisme, la France a le plus haut taux de croissance de la zone euro, son taux de chômage est au plus bas depuis à peu près quinze

Détaillé quant à ses objectifs de gains de productivité et de calendrier, le projet ne formulait initialement aucun objectif précis d'amélioration de la qualité du service rendu aux usagers. Érigé en emblème de la logique de modernisation et de simplification des démarches administratives, ce plan révèle les manquements des intentions des réformateurs de l'État,

par les centres d'expertise et de ressources des titres (CERT), qui mettent en oeuvre, non sans difficulté, la dématérialisation de la délivrance des quelque 24 millions de titres tels que les passeports, les permis de conduire ou les cartes grises.

On y compte jusqu'à 30 % de contractuels, qui se substituent aux titulaires. Les points de contact, heureusement, subsistent, et ils sont le signe que l'ambition portée par les téléprocédures n'est pas satisfaisante pour les personnes fragiles et dépendantes. Cette déshumanisation du rapport des citoyens à l'État et à ses agents, loin de générer des économies, engendre un surcoût de 15 millions d'euros par an pour l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et de 40 millions d'euros en outils informatiques, quand vous supprimez 1 000 postes.

entre avril 2020 et septembre 2021. Il faut conclure. En l'absence d'alternative, ces publics potentiellement éloignés de la langue française et du numérique risquent, faute d'accueil, d'être privés de leurs droits et placés en situation d'illégalité.

de bonne gestion. Et cela doit s'accompagner d'un exercice de pédagogie. Bien entendu, et je me permets là une adresse à la Haute Assemblée, quand